La séance est ouverte. Le compte rendu intégral de la séance du jeudi 23 septembre 2021 a été publié sur le site internet du Sénat. Il n'y a pas d'observation ? ... Le procès-verbal est adopté. est adopté. J'ai le regret de vous faire part du décès de notre ancienne collègue Kheira Bouabsa, qui fut sénateur de la Communauté de 1959 à 1961.

du citoyen : « Tous les Citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique [ ...]. » À l'occasion de cet anniversaire, nous pouvons en saluer les fondateurs Alain Lambert et Didier Migaud, qui ont grandement contribué, par leurs travaux et leur détermination, à améliorer notre architecture budgétaire.

que ce soit essentiel pour faire la transparence sur l'usage de la contribution publique. Par ailleurs, le Parlement vote la totalité des crédits de chaque mission budgétaire, ce qui n'était pas non plus le cas avant la LOLF, car, je le rappelle, les crédits de l'année précédente étaient simplement reconduits par un vote unique.

en autorisant le dépôt d'amendements parlementaires visant à modifier les moyens alloués aux programmes budgétaires, alors que le dépôt de tels amendements était tout bonnement impossible par le passé. Il s'agit aussi d'une réussite en ce qui concerne la performance de la dépense publique. Les progrès apportés par ce texte sont à cet égard indéniables.

d'un moyen concret donné au Parlement en matière de contrôle budgétaire, ce qui contribue aussi à la démocratisation de l'information en matière de finances publiques. Pour autant, malgré ces succès et ces avancées, la pratique n'a pas épuisé l'ensemble du potentiel de la LOLF. Nous devons nous saisir des moyens qu'elle met à notre disposition.

pour que la justification au premier euro remplace vraiment la discussion sur les seules mesures nouvelles, à la fois au Parlement et au sein des administrations. Nous ne devons pas tomber dans le piège de la « bureaucratisation de la réforme » sur laquelle nous alertaient Alain Lambert et Didier Migaud dès 2006.

C'est la volonté exprimée par les députés Laurent Saint-Martin et Éric Woerth, auteurs de cette proposition de loi organique et, par ailleurs, respectivement rapporteur général et président de la commission des finances de l'Assemblée nationale. Je tiens à les remercier devant vous pour la qualité de leurs travaux, et remercier l'ensemble des parlementaires qui y ont contribué.

Qu'il s'agisse de la commission sur l'avenir des finances publiques présidée par Jean Arthuis, ou de la Cour des comptes, le constat dressé est similaire : pour assainir les finances publiques, la programmation pluriannuelle des budgets doit impérativement être renforcée, objectif auquel je souscris sans réserve. La proposition de loi organique prévoit d'instaurer une règle en matière de dépenses qui nous permettra de nous inscrire encore davantage dans une maîtrise pluriannuelle de nos finances publiques. Cet objectif d'évolution des dépenses est d'autant plus important que le Gouvernement pourra compter sur la vigilance du Haut Conseil des finances publiques (HCFP) pour détecter les écarts entre ce qui était prévu et ce qui a été fait.

C'est une volonté forte, qui rejoint tout à fait la ligne que nous nous sommes fixée : amorcer la décrue de notre dette dans les années à venir, objectif qui sera atteint notamment si l'on suit de manière précise les conditions de sa gestion.

mesure va dans le sens d'un cycle budgétaire plus transparent, objectif auquel le Gouvernement est particulièrement attaché. La proposition de loi organique prévoit également un contrôle du HCFP sur la compatibilité des dispositions des projets de loi de programmation sectorielle avec celles de la loi de programmation des finances publiques c'est une disposition que nous soutenons, dans la mesure où elle est indéniablement au service de la sincérité budgétaire. Il s'agit d'asseoir la crédibilité des lois de programmation des finances publiques en évitant que d'autres lois de programmation n'en fragilisent le respect et de garantir les moyens dont l'État dispose pour la mise en oeuvre des lois de programmation sectorielle.

La sincérité budgétaire n'a de sens que si les lois financières sont compréhensibles : il s'agit d'un enjeu démocratique. Les auteurs de la présente proposition de loi organique ont donc pour ambition de réorganiser la présentation des lois de finances en vue d'en améliorer la lisibilité et la transparence

Dans son rapport d'information, Alain Lambert résumait ainsi l'esprit de cette loi : « Le contrôle parlementaire sur les finances publiques est une ardente obligation sans laquelle les fonctions du Parlement ne sauraient être réellement exercées.

». La proposition de loi organique améliore également le processus législatif. De fait, le renforcement des pouvoirs du Parlement passe aussi par une réorganisation du calendrier législatif. S'agissant du cadrage général, le débat d'orientation des finances publiques serait refondé s'y substituerait une obligation pour le Gouvernement de fournir au Parlement les plafonds de crédits par mission avant le 15 juillet. Aussi y aurait-il un débat unique portant à la fois sur l'orientation des finances publiques au moment de la présentation du programme de stabilité, au mois d'avril, et sur ce programme de stabilité. Dans la même logique, le décalage au 1 mai de la date limite de dépôt du projet de loi de règlement entérinerait la pratique actuelle pour laisser davantage de temps au Parlement de mener ses travaux d'évaluation. Enfin, le texte que vous vous apprêtez à discuter a été enrichi par votre commission des finances.

ou encore à décorréler la date de remise au Parlement des projets annuels de performance et des annexes générales pour permettre à celles-ci d'être les plus complètes possible. Mesdames, messieurs les sénateurs, cette proposition de loi organique contribue à doter l'État d'outils rénovés, précieux pour le Parlement comme pour le Gouvernement.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous voici réunis pour examiner deux propositions de loi qui visent principalement à réformer la loi organique relative aux lois de finances, ans après son adoption. Nous devons le faire d'une « main tremblante », car il s'agit, ni plus ni moins, de notre « constitution financière ». Permettez-moi d'abord de saluer le travail de nos collègues députés à l'origine de ces textes, en particulier

Pour autant, l'examen de ces textes par notre assemblée nous paraît intervenir à contretemps. Bien sûr, il est plus que temps de s'intéresser- pour le souhaiter -au retour à une situation budgétaire plus saine. Cela fait des années que le Sénat rappelle aux gouvernements successifs la nécessité de retrouver un niveau moins élevé de prélèvements obligatoires, de réduire le déficit et, surtout, de maîtriser la dépense publique. La crise sanitaire ne justifie pas à elle seule les errements en la matière. pour examiner ces propositions de loi se situe en pleine sortie de crise sanitaire et économique, à presque six mois des élections présidentielle et législatives. Disons-le tout net, nous ne sommes pas dupes ! Sous couvert d'un travail sérieux réalisé par nos collègues députés il y a maintenant près de deux ans, la majorité gouvernementale en profite, alors que les vannes sont manifestement encore grandes ouvertes dans le cadre du pour donner une impression de sérieux budgétaire à nos partenaires européens. Ces propositions de loi, qui visent notamment à inscrire un objectif pluriannuel de dépenses des administrations publiques, comme vous venez de le rappeler, monsieur le ministre, ne s'appliqueront que plus tard, après les séquences électorales alors que mille et une promesses budgétaires auront été faites par le président sortant. Il suffit pour s'en convaincre de lire la presse au gré des visites présidentielles et/ou ministérielles, et d'observer l'augmentation de la quasi-totalité des crédits des missions du prochain projet de loi de finances. Ces propositions de loi arrivent donc trop tard, mais peut-être aussi trop tôt, puisqu'une réforme du pacte de stabilité pourrait aboutir au niveau européen d'ici à 2022, ce qui conduirait à modifier profondément la programmation pluriannuelle.

la commission des finances souscrit à nombre d'entre elles, au premier rang desquelles la fixation d'une norme pluriannuelle de dépenses des administrations publiques. La maîtrise de la dépense publique est indispensable si l'on veut retrouver un souffle budgétaire. Nous proposons toutefois, dans le prolongement des conclusions de la commission Arthuis, que soient identifiées les dépenses d'avenir, afin que les mesures contribuant à une croissance économique de long terme, ainsi qu'au progrès social et écologique ne soient pas sacrifiées. Nous souhaitons également que les lois de programmation des finances publiques puissent être plus aisément révisées lorsque leurs orientations pluriannuelles sont manifestement dépassées. Le Gouvernement n'a pas jugé utile de le faire alors que, depuis la crise des « gilets jaunes », l'actuelle loi de programmation des finances publiques n'a plus ni portée ni consistance. Nous pensons également que le Haut Conseil des finances publiques doit pleinement jouer son rôle. Nous proposons de lui confier le soin de s'assurer de la « cohérence »- plutôt que du « réalisme », comme vous l'avez expliqué, monsieur le ministre -des prévisions budgétaires au regard notamment des données macroéconomiques. La proposition de loi organique améliore l'examen de la loi de finances et le calendrier budgétaire. Je salue la simplification apportée, puisque le texte prévoit l'examen de l'ensemble des recettes en première partie. Nous proposerons d'aller plus loin s'agissant des taxes affectées. Le débat unique en avril, qui regroupe à la fois le débat sur le programme de stabilité et le débat d'orientation des finances publiques, est également bienvenu : nous pensons que c'est à ce moment-là que le rapport sur la dette doit être remis. Nous profitons de ces textes pour mieux encadrer l'exécution budgétaire et renforcer le contrôle et l'information du Parlement, notamment sur les reports de crédits. Nous souhaitons ainsi améliorer l'accès aux données.

placer au coeur du débat budgétaire la question des dépenses publiques et de la dette ; enfin, « toiletter » la LOLF, vingt ans après son adoption. Je commencerai par ce dernier point : nous approuvons les dispositions visant à réviser les modalités d'examen de la loi de finances. Ainsi en est-il du resserrement des collectifs budgétaires de fin d'année sur les seuls mouvements de crédits. Nous souscrivons aussi à l'idée de discuter de l'ensemble des recettes en première partie de la loi de finances. Nous proposons d'aller plus loin : pour que le Gouvernement respecte davantage l'autorisation budgétaire,

de la possibilité de prendre des mesures affectant uniquement des années ultérieures à l'exercice à venir, la ratification des conventions internationales en matière fiscale, ou encore la restriction des questionnaires budgétaires.

La dépense publique est une question centrale, à laquelle la commission des finances prête toute l'attention nécessaire, mais focaliser le débat public sur le seul niveau de cette dépense sans considération de sa qualité nous apparaît particulièrement réducteur. La commission Arthuis avait certes proposé de définir un objectif en matière de dépenses, mais elle avait aussi demandé de fixer « un périmètre et un niveau plancher de dépenses d'avenir » en début de mandature pour que cette maîtrise des dépenses ne se fasse pas- comme par le passé -au détriment des dépenses favorables à la croissance. Elle citait les dépenses vertes, les dépenses d'investissement et d'innovation et celles qui sont favorables au capital humain.

De même, nous considérons qu'un budget, ce sont des dépenses, mais aussi des recettes, et que l'on ne peut pas appeler l'attention que sur une seule de ces deux composantes. Je ne reviendrai pas sur ce que je pense des allégements de fiscalité sur les entreprises ou le patrimoine, tout particulièrement en période de récession. Le débat politique doit avoir lieu, car le « désarmement fiscal » auquel nous avons assisté est un facteur important de déséquilibre de nos comptes publics. Il est à noter que le rapport Arthuis chiffre à 50 milliards d'euros l'effort à faire porter sur nos dépenses, quand le Gouvernement se félicite d'une baisse d'impôt de ... 50 milliards d'euros- -durant ce quinquennat, baisse que l'on retrouve aujourd'hui dans la dette. Chacun sait que notre dette publique n'a cessé d'augmenter : elle atteint désormais 115 % du PIB. Notre commission a tenu une table ronde sur ces sujets, alors qu'un débat en séance publique a également eu lieu. À chaque examen d'un texte financier, nous en discutons. C'est pourquoi, à titre personnel, je pense que rien n'impose d'ajouter un débat annuel sur la dette dans la loi organique. Chaque assemblée peut et doit rester maîtresse de son ordre du jour. sur la question de la programmation. Nous appelons tous de nos voeux une programmation réaliste de nos finances publiques et le respect de ce principe. La loi de programmation adoptée en début de quinquennat est devenue obsolète dès la fin de et les mesures prises pour répondre- très justement -au mouvement des « gilets jaunes ». Malgré nos demandes réitérées, le Gouvernement s'est toujours refusé à la modifier, si bien que, cette année, notre dette publique est supérieure de 20 points à l'objectif toujours en vigueur. Aucune révision des contrats de Cahors pour les collectivités locales n'a non plus eu lieu, l'application de la loi étant seulement « suspendue ». Dire que le prochain quinquennat permettra de respecter les engagements pris c'est faire le pari d'une autre gouvernance que celle que nous avons actuellement. Les textes dont nous discutons aujourd'hui ont vocation à renforcer la maîtrise de la dépense publique et l'information du Parlement,

La vertu appartiendra donc au prochain quinquennat. En résumé, à l'avenir, nos finances publiques ne devront rien à cette modification de notre cadre organique, mais tout à la seule volonté politique des majorités démocratiquement élues ! Bravo ! La parole

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous examinons cet après-midi deux textes distincts, mais qui visent un même objectif : modifier le cadre dans lequel le Parlement vote le budget. ans après l'adoption de la loi organique relative aux lois de finances, cet exercice est le bienvenu. S'agit-il d'une révolution ? Non, certainement pas. S'agit-il d'une révolte ? Même pas. Il s'agit ni plus ni moins d'une réforme technique et méthodique, pour ne pas dire un peu ésotérique. Soyons clairs : il faut être rompu à l'exercice des examens budgétaires pour comprendre l'utilité de ces textes ... Mais comme les Français sont plus doués pour faire la révolution que les réformes, pour reprendre la formule de Tocqueville,

Elle a permis de mieux encadrer les discussions, de clarifier la présentation du budget et de renforcer le rôle du Parlement dans sa mission de contrôle. Cependant, vingt ans après, nous avons identifié les défauts et les lacunes de ce grand texte, qui ne pouvait pas être parfait. Des ajustements s'imposent, et nous allons pouvoir en débattre sereinement. En l'occurrence, mieux vaut de petits ajustements qu'un grand chambardement.

Sans doute, car l'un n'empêche pas l'autre. Le moment est toujours le bon quand il s'agit de renforcer l'efficacité de l'action publique. De fait, ces deux textes nous permettront de voter des budgets plus sincères dans des conditions plus sereines. Ils vont donc tous deux dans le bon sens.

ce sujet. Nous sommes tous d'accord ici pour dire que cet exercice démocratique est sain, pour la simple et bonne raison que nous ne sommes pas d'accord sur le fond. Grâce à ce texte, nous pourrons peaufiner nos diagnostics et faire valoir nos orientations politiques. En clair, nous serons dans notre rôle. Il en va de même de la révision du calendrier budgétaire. La proposition de loi organique consacre, dans la LOLF, plusieurs des bonnes pratiques mises en place par le Gouvernement avant la pandémie. la création d'une nouvelle catégorie de lois de finances pérennisera les bonnes habitudes que nous avions prises avant la crise. Il s'agit de concentrer l'essentiel des mesures fiscales et budgétaires durant l'automne. Je crois que cette pratique donnera davantage de lisibilité et de sécurité aux Français. Il en va de même de la distinction entre dépenses de fonctionnement et dépenses d'investissement dans les documents budgétaires. Nous avons été nombreux au sein de cet hémicycle à dire que l'endettement public ne devait pas servir à financer des dépenses de fonctionnement. Cette distinction est donc la bienvenue, et c'est à mes yeux l'un des points forts de ce texte. Sur ce point, prenons garde de ne pas faire de mauvais procès. Distinguer, ce n'est pas discriminer. Identifier, ce n'est pas hiérarchiser. On peut distinguer deux catégories sans forcément considérer par la même occasion que l'une est utile, et l'autre non. La justice, la police et l'armée relèvent du fonctionnement davantage que de l'investissement : elles sont pourtant essentielles. Distinguer entre fonctionnement et investissement est une pratique normale dans nos collectivités locales. Pour une fois que nous pouvons améliorer les débats parlementaires en nous inspirant de la démocratie locale, nous ferions mieux de nous en réjouir. Il est primordial de mieux identifier les dépenses qui préparent l'avenir et celles qui relèvent de la gestion courante. En vérité, ce devrait être notre unique obsession

d'ailleurs, le principe d'annualité budgétaire, de valeur constitutionnelle, garantit cette faculté au Parlement -, mais il est urgent que nous reprenions le contrôle de nos finances publiques. Le Gouvernement comme le Parlement doivent prendre des engagements forts pour réduire l'endettement public. Les propositions que nous allons examiner n'y suffiront certes pas, mais elles y contribueront utilement. Pour l'essentiel, les débats se poursuivront dans quelques semaines dans le cadre de

Monsieur le président, monsieur le ministre,

Néanmoins, le groupe RDPI et moi-même regrettons le refus du Sénat de s'associer depuis le départ à ce travail, avec le Printemps de l'évaluation pourtant engagé. Je souhaite rappeler l'esprit de consensus qui devrait être le nôtre en matière de gestion et d'organisation des finances publiques, car consensus il y a eu par le passé ... Promulguée le 1 août 2001, la LOLF a profondément transformé l'architecture budgétaire de l'État, permettant un meilleur suivi

textes examinés aujourd'hui. Cela étant, notre groupe a quelques points de désaccord avec la position des rapporteurs. Par conséquent, je souhaite attirer votre attention sur les deux amendements que je défendrai au nom du groupe RDPI. Le premier concerne l'introduction de la référence aux « dépenses d'avenir » comme indicateur spécifique en loi de programmation des finances publiques. L'amendement que je présenterai vise à revenir à la rédaction de l'article 1 de la proposition de

il a donc pour vocation non à distinguer les dépenses d'avenir et les dépenses de fonctionnement, mais à présenter une vision consolidée de l'évolution des dépenses par rapport à la programmation. Nos débats en commission l'ont bien rappelé ! Nous avons l'occasion de doter la LOLF de nouveaux outils performants. J'ose espérer qu'il puisse être question d'outils neutres et transpartisans. la notion de « dépenses d'avenir » n'est pas définie avec clarté et ferait, à n'en pas douter, l'objet d'instrumentalisations politiques de toutes parts. Je crois d'ailleurs que ce n'est pas au Gouvernement d'évaluer la qualité de ses propres investissements en construisant un tel indicateur, qui se révélerait à l'usage particulièrement arbitraire. C'est au Parlement et à la représentation nationale d'endosser ce rôle dans le cadre de ses travaux d'évaluation et de contrôle. Le second amendement a pour objet de supprimer, à l'article 12 de la proposition de loi organique, la possibilité pour le Haut Conseil des finances publiques d'émettre un avis sur l'exécution de l'année en cours, lorsqu'il est saisi à l'occasion du projet de loi de finances. Nous estimons que le contrôle de l'exécution doit être effectué par le Haut Conseil une fois l'exercice clos, et non en cours d'exercice. Cela permettrait de maintenir un équilibre sain entre la liberté d'action du Gouvernement et le contrôle par le Parlement sans que le Haut Conseil soit amené à se prononcer en cours d'exercice autrement que lors du dépôt d'un projet de loi de finances rectificative, comme c'est le cas aujourd'hui. Tels sont les deux amendements que je défendrai après la discussion générale. Mes chers collègues, au-delà de ces deux points, je crois que nous sommes face à une occasion que nous devons saisir. Plus que jamais, nous devons réformer la gouvernance de nos finances publiques et moderniser notre approche. Réformer le calendrier budgétaire et la procédure d'examen des textes financiers pour améliorer la lisibilité des lois de finances et l'articulation avec la programmation pluriannuelle ; renforcer la portée de l'autorisation budgétaire en limitant notamment le recours aux taxes affectées aux taxes affectées ; retrouver l'esprit de la LOLF en renouvelant la démarche de performance et la culture du résultat ; consolider l'information du Parlement, ainsi que les pouvoirs d'évaluation et de contrôle de la commission des finances, afin de rendre possible un véritable « " chaînage vertueux " entre l'évaluation des résultats passés, l'autorisation

J'écoutais avec attention l'actuel président du Haut Conseil des finances publiques, Pierre Moscovici, lors de son audition la semaine dernière par la commission des finances, à l'occasion de la présentation de son avis sur le projet de loi de finances pour 2022. Je dois dire que j'ai été plutôt convaincu. Convaincu par son propos et et son appel à saisir l'occasion de l'examen en séance publique pour faire avancer les choses, dans l'intérêt des finances publiques de la France et dans l'intérêt général. J'ai été convaincu également par sa volonté de nous alerter sur la gestion à long terme de notre endettement actuel. Le Gouvernement a pris les mesures nécessaires et la stratégie du « quoi qu'il en coûte » a démontré son efficacité. Néanmoins, la question de l'endettement se posera encore sans doute pendant de nombreuses années et nous devons nous doter des outils permettant d'y répondre. Ce sont autant de raisons pour lesquelles le groupe RDPI votera pour l'adoption de ces textes.

comme un bonheur n'arrive jamais seul, nous entamons cette rentrée budgétaire avec deux propositions de loi qui s'attellent à un sujet relativement technique : la modernisation du cadre des lois de finances. Au risque de rappeler une évidence, c'est la raison d'être du Parlement depuis plus de deux cents ans que d'examiner le budget des pouvoirs publics et d'autoriser à la fois les prélèvements obligatoires et les dépenses des administrations. L'article XIV de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen énonce que « tous les Citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique nécessité de la contribution publique [ ...] ». Les lois de finances diffèrent des autres lois ordinaires à la fois par leur contenu, fait de nombreuses données chiffrées, et par leur procédure d'examen, qui obéit à des délais constitutionnels stricts, ainsi qu'à des règles de recevabilité financière et organique non moins contraignantes. Les difficultés inhérentes à l'examen des lois de finances sont connues : lourdeur et complexité de la phase du projet de loi de finances initial à l'automne ; au contraire, pauvreté de l'examen du projet de loi de règlement et du débat d'orientation des finances publiques au début de l'été contrôle insuffisant de l'exécution. Ainsi, la prévision initiale est toujours frappée d'incertitudes et il n'existe pas de budget dont l'exécution corresponde exactement à la loi initialement adoptée. L'enjeu est donc de voter des prévisions de recettes et de dépenses à la fois crédibles et sincères. Une autre critique formulée depuis longtemps à l'encontre de la LOLF la mise en place d'une comptabilité d'État véritablement moderne et l'instauration d'une culture du résultat qui permette une amélioration de la qualité de la dépense publique. Il faut se souvenir de l'ampleur du travail réalisé à l'époque de la rédaction de la LOLF. L'État s'était alors doté d'un cadre réellement nouveau pour ses finances, par rapport à l'ordonnance organique de 1959- un cadre d'une grande complexité néanmoins, surtout comparé à celui de la gestion des finances locales, et qui n'a pas permis une amélioration de la situation des finances publiques. Certes, les prérogatives du Parlement ont été renforcées : l'information budgétaire est relativement abondante- au point que l'on s'y perd parfois -et l'on examine et vote les crédits programme par programme, mission par mission, un niveau de détail qui n'existait pas avant 2005. Toutefois, au-delà du cadre organique, nous aurons toujours les contraintes de recevabilité des amendements liées à l'article 40 de la Constitution et à l'application qui en est faite : les parlementaires ne peuvent pas compenser une charge publique et toute baisse de recette doit être compensée par une recette équivalente. C'est peut-être une sécurité pour les finances publiques, mais qui se paye par des marges de manoeuvre très restreintes pour les parlementaires, souvent réduits à approuver ou rejeter le budget ou les amendements proposés par le Gouvernement, sans pouvoir, eux-mêmes, amender significativement Enfin, notre cadre budgétaire est aujourd'hui fortement influencé par les règles en vigueur au niveau européen : depuis le traité de Maastricht, l'adoption du pacte de stabilité et de croissance et, en 2012, le traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance- dont la création du Haut Conseil des finances publiques est une conséquence -, le Gouvernement doit transmettre à la Commission européenne des engagements budgétaires clairs et argumentés. Le temps n'est pas si loin où la France faisait encore l'objet d'une procédure pour déficit excessif. sans représenter un big-bang budgétaire, les deux textes que nous examinons apportent des améliorations et des clarifications utiles, ainsi qu'une occasion de débattre sur le fond des règles budgétaires. Parmi les améliorations, je relève la doctrine d'emploi des ressources affectées, qui donne souvent lieu à des difficultés d'interprétation lors de l'examen des Le Gouvernement inscrit également dans le marbre le principe de la loi rectificative de fin de gestion, pratique instaurée depuis le début de ce quinquennat. On peut néanmoins regretter que la commission des finances ait supprimé certaines dispositions, comme la consécration de l'évaluation de l'impact environnemental des dépenses publiques, improprement appelée « budget vert ». Pour ces différentes raisons, les membres du groupe du RDSE devraient voter majoritairement pour l'adoption de ces deux propositions de loi.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, moderniser la gouvernance des finances publiques est un projet ambitieux, tout comme vouloir rendre plus lisibles la dépense, l'impôt et la taxe,

il ne trouve presque aucun débouché dans ces textes. Nous nous sommes posé deux questions. Comment, grâce à ces propositions de loi, les citoyens amélioreront-ils leur compréhension des débats budgétaires et se les approprieront-ils

puisque la LOLF est confortée dans ses principes et ses objectifs. Je dirai, monsieur le ministre, que vous appliquez aux mêmes causes les mêmes remèdes. Sur ce point, nous sommes force de proposition laisser les parlementaires soumettre au débat un contre-budget, sans dépasser le montant global des crédits, de sorte que personne, pas même le Gouvernement, puisse nous qualifier de dépensiers. Nous vous présenterons ce que nous ferions si nous assumions la responsabilité

un plan de relance sans planification est synonyme de tout-venant et de débudgétisation des crédits traditionnels ... Cette modernité dont vous vous prévalez est, à nos yeux, un concept assez creux. La logique de performance et de gestion induite par la LOLF perdurera au détriment de la qualité du débat et de la décision budgétaire. Vous confortez notre impuissance- certains pourraient parler d'allégeance -face à la Commission européenne et aux traités européens. La loi de programmation des finances publiques devrait-elle être conforme aux traités européens ?

Voilà un cap et une utilité restaurée des lois de programmation ! Tout le contraire d'une « modernité » qui choisit d'imposer les mécanismes de réduction des dépenses publiques, chers à la Commission européenne, une modernité bien loin d'être source de changement- c'est la conception qui préside à tous les choix budgétaires depuis plusieurs décennies et, plus encore, depuis l'avènement de la LOLF. Notre groupe propose une autre solution : rompre avec cette logique budgétaire, que nous qualifions de « dangereuse

Des services se retrouvent avec l'interdiction de recruter un fonctionnaire, mais avec assez d'argent pour faire un chèque deux fois plus élevé à des cabinets privés. On appelle cela la « maîtrise des dépenses » Les effets des politiques soumises à ces cadres budgétaires sont « antisociaux » et contre-productifs. La logique de performance de la LOLF fait donc bel et bien figure de mythe. Votre seule réponse à tous ces maux et au déclin des marges de manoeuvre du Parlement et des groupes politiques dans l'élaboration du budget, c'est de rajouter du papier à destination des parlementaires et des citoyens

Il faut réformer la LOLF pour raffermir la démocratie budgétaire. C'est le sens de notre action, et de notre opposition à ces propositions de loi. La parole est à M. Vincent

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, quelle est notre ambition à travers ces textes ? Nous essayons de tirer les conséquences d'un certain nombre de difficultés rencontrées dans l'application de la LOLF.

Le lien avec la loi de programmation des finances publiques est aussi renforcé, grâce à un compteur des écarts. La commission a posé la question, légitime, de l'équilibre entre ces innovations procédurales et le respect des droits du Parlement. Elle a introduit dans le débat une définition plutôt large

Le groupe Union Centriste plaide depuis longtemps pour un renforcement de la maîtrise de nos dépenses publiques. Nous accueillons ainsi favorablement les modifications apportées au cadre pluriannuel des finances publiques. Certes, la volonté politique primera toujours en ce domaine. Il n'empêche que les règles budgétaires sont utiles et nécessaires pour donner des points de repère. Dans la même optique, nous nous félicitons de la création d'un débat sur la dette publique et sa soutenabilité. Notre collègue Vincent Delahaye défendra un amendement, visant à préciser le contenu du rapport relatif à la dette publique. Je me réjouis de l'adoption par notre commission de l'amendement de notre collègue Sylvie Vermeillet, prévoyant la remise, parmi les annexes au projet de loi de règlement, de tableaux récapitulant le nombre d'emplois rémunérés par l'État, ainsi que sa variation. Le nombre d'agents publics a augmenté à un rythme deux fois supérieur à celui de la population depuis le début des années 1980. En tant que rapporteur spécial du budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » (Bacea), j'ai bien sûr porté une attention toute particulière à l'article 4 de la proposition de loi organique, tendant à modifier les règles relatives aux budgets annexes. La commission a adopté l'amendement que j'ai déposé sur ce point, et je remercie nos deux rapporteurs de leur attention vigilante et de leur soutien. À la suite d'un travail approfondi avec les différents acteurs du secteur du contrôle aérien, notamment les administrations et votre ministère, monsieur le ministre, j'ai souhaité rectifier le dispositif adopté par l'Assemblée nationale afin de clarifier le périmètre des opérations retracées-

ou une moindre incitation à aller de l'avant en matière de performances. Évidemment, il faut un régulateur fort, et nous aurons l'occasion de revenir sur ce point. Nous clarifions également les notions de ressources et de charges des budgets annexes, en les alignant sur les définitions prévues aux articles 3, 5 et 25 de la LOLF. Mes chers collègues, le renforcement de la maîtrise de nos dépenses publiques dans les discussions budgétaires est un sujet de préoccupation pour tout le monde- en tout cas pour les membres du groupe Union Centriste. Considérant que ces deux textes vont dans le bon sens, et malgré certains points d'amélioration restant en suspens, ceux-ci voteront pour l'adoption de ces deux propositions de loi.

améliorer l'information du Parlement sur les finances publiques et réorganiser la discussion parlementaire des lois financières pour en assurer une meilleure visibilité, tels sont les objectifs affichés par la proposition de loi organique et la proposition de loi mises en débat, aujourd'hui,

Certes, nous ne pouvons qu'approuver la volonté de réorganisation, souhaitant nous aussi éviter la répétition de débats quasi identiques en première et seconde parties du budget.

J'ajoute que la portée des dispositions visant à contrôler la dépense publique reste limitée, les lois de programmation pluriannuelle n'ayant aucune autorité sur les lois de finances annuelles. Le Parlement peut très bien établir une programmation sur plusieurs années et voter, l'année suivante, un budget en contradiction totale

de possibilités de recours à des organismes extérieurs en temps voulu ou aux administrations publiques concernées par le biais de questionnaires budgétaires, par exemple. indispensable de renforcer l'évaluation chiffrée des incidences des dispositions introduites par le Gouvernement en cours d'examen du projet de loi de finances, comme la LOLF le prévoit aujourd'hui pour les dispositions initiales du projet de loi de finances affectant les ressources ou les charges de l'État. Par ailleurs, l'ambition de la LOLF était de mesurer l'écart pouvant exister entre les objectifs affichés et les effets concrets de la mise en oeuvre d'une politique.

Cela serait pourtant nécessaire pour renforcer les pouvoirs de contrôle du Parlement. En effet, si le texte que nous étudions aujourd'hui prévoit déjà, et c'est une avancée, une information plus formalisée sur les écarts entre crédits votés et crédits réalisés, cela reste un bien petit pas.

renforcement de l'évaluation des dépenses fiscales- sans pour autant nier leur utilité -, mise en perspective de la trajectoire des recettes, afin de ne pas limiter le débat à la seule et unique question de la dette. En effet, si rien dans ce texte ne vient imposer une « règle d'or », l'approche par la limitation de la dépense publique et la mise en avant du seul enjeu de la dette imprègnent son esprit et, très largement, nos débats. l'enjeu devrait être bien plus global ; il concerne aussi les recettes de l'État. Quel niveau de fiscalité ? Pesant sur qui ? Évoluant comment ? Et pour répondre à quels besoins ? Comment parler de dépense et de dette publiques sans parler d'investissement et de services publics, de transition écologique, d'investissements d'avenir ? Sur ces sujets,

du pilotage pluriannuel des finances publiques apparaît décevant, dans la mesure où les objectifs fixés par les lois de programmation ont rarement été atteints. » Elle indiquait également que « la fragmentation du cadre de la dépense publique nuit à la clarté des choix et à la bonne compréhension de l'usage des deniers publics Cette proposition de loi se veut une tentative de réponse à ces critiques. En juin dernier, sur l'initiative du groupe CRCE, le Sénat a débattu du rôle du Parlement dans l'élaboration des lois de finances. À cette occasion,

Par exemple, ne faudrait-il pas imposer à l'État les mêmes règles qu'aux collectivités territoriales : présenter une section de fonctionnement équilibrée, encadrer l'évolution des dépenses de fonctionnement, limiter la possibilité de recourir à l'endettement pour financer l'investissement,

Toutefois, ce texte ne doit pas être l'occasion de dessaisir le Parlement de ses prérogatives au bénéfice d'organismes extérieurs. Les sénateurs comme les députés ont toute légitimité pour réaliser les chiffrages des différentes mesures, à condition bien entendu que l'ensemble de l'information soit transparente. Fort de son regard objectif, le Haut Conseil des finances publiques (HCFP) doit venir en appui des investigations parlementaires. Il ne doit pas remplacer le Parlement. Il veillera notamment au respect des objectifs pluriannuels de réduction des dépenses et devra pouvoir obtenir du Gouvernement une justification des écarts observés par rapport à la cible pluriannuelle.

Il aurait certainement été plus efficient d'actualiser la loi de programmation des finances publiques, obsolète depuis plusieurs exercices budgétaires, et de consacrer tous nos efforts aux échanges européens. À cet égard, la taxonomie verte En effet, rien ne sert de sanctuariser la pratique du budget vert, avec une présentation annuelle au Parlement des conséquences environnementales du projet de loi de finances, si dans le même temps, au niveau de l'Union européenne, on refuse de considérer comme vertes des dépenses en faveur d'une énergie totalement décarbonée.

en confiant aux parlementaires un pouvoir de contrôle sur l'exécution des lois de finances. Aujourd'hui, vingt ans après l'adoption de ce texte, il était sans doute logique de considérer qu'une évolution était nécessaire. Pour autant, la proposition de loi organique qui nous est soumise ne nous permet pas d'afficher une satisfaction sans faille.

cette proposition de loi organique interroge : soit elle arrive trop tard, à l'issue d'un quinquennat au cours duquel aucune velléité de réforme n'a réellement émergé arrive trop tôt, alors que les effets de la crise sanitaire sur l'économie et les finances publiques ne sont pas encore tous connus et qu'une réforme du pacte de stabilité et de croissance européen pourrait être à l'ordre du jour des prochains mois. Ce texte, dont le contenu demeure tout de même assez technique, n'en cache pas moins une approche très politique des finances publiques. En focalisant le débat sur la dette, il oriente de fait les discussions. s'agit évidemment d'un sujet d'importance : aggravée par la crise sanitaire, la dette nécessite une attention particulière. Elle ne saurait toutefois être la boussole qui détermine le cap à donner aux politiques publiques. Si la crise sanitaire a accru la dette, elle a permis de relativiser la perception que nous en avons. Une fois dépassée, la ligne rouge des 100 % du PIB, réputée infranchissable, pourrait ainsi conduire à une autre réflexion sur les finances publiques. Les politiques publiques sont les grandes oubliées de cette réforme de la LOLF. Ce sont pourtant elles qui nous réunissent tous ici et qui nourrissent nos discussions.

Nous le voyons bien : les orientations des finances publiques doivent découler des politiques publiques, et non l'inverse. Au lieu de cela, l'orthodoxie budgétaire est une nouvelle fois de mise, au nom d'une doctrine libérale annonciatrice de réformes où la justice sociale n'aura guère sa place. cette proposition de loi organique présente également de nombreux aspects techniques ne posant pas de difficulté particulière. Ainsi, la présentation du budget en dépenses d'investissement et de fonctionnement facilitera sa compréhension et son analyse. De plus, l'utilisation et l'évaluation du prélèvement sur recettes à destination des collectivités territoriales pourraient ouvrir la voie à un débat politique fort, à la hauteur des enjeux financiers des communes, des départements et des régions. Néanmoins, la volonté affichée d'une meilleure information parlementaire et d'une simplification de la procédure peine à atteindre son but. S'il n'est pas certain que les débats budgétaires soient plus lisibles une fois ce texte adopté, l'orientation politique annoncée, elle, est parfaitement claire.

vont soutenir ces deux propositions de loi, organique et ordinaire, qui, globalement, améliorent le cadre de fonctionnement de la gouvernance financière publique.

d'apports méritent d'être soulignés, notamment pour les finances publiques locales. L'organisation, en amont de la discussion du projet de loi de finances, d'un débat sur la situation des finances des collectivités territoriales constitue assurément une mesure opportune. Nous espérons que les apports de la commission des finances quant au contenu du rapport prévu à cet effet seront conservés à l'issue de la CMP. Je pense, en particulier, à l'évolution des charges résultant des transferts de compétences ainsi qu'à l'information du Parlement sur l'efficacité des transferts financiers entre l'État et les collectivités territoriales. Plus généralement, la consolidation de la pluriannualité budgétaire devrait opportunément renforcer la démarche de performance et la logique de résultat qui sont à l'origine de la LOLF.

relevé -, les lois de programmation des finances publiques peuvent être remises en cause chaque année, alors qu'elles devraient contraindre le Gouvernement et le Parlement à proposer et à voter des lois cohérentes avec elles, notamment les lois de finances annuelles. Or la valeur constitutionnelle reconnue au principe d'annualité budgétaire prive les lois pluriannuelles de programmation des finances publiques d'une autorité juridique supérieure à celle des lois de finances. Le Gouvernement et le Parlement pourront toujours adopter des dispositions contraires contraires aux règles budgétaires inscrites dans les lois de programmation, notamment les règles d'évolution des dépenses publiques comme les normes dites « en valeur » et « en volume ». Un cadre budgétaire est certes nécessaire pour obliger le Gouvernement à s'expliquer lorsque des comités budgétaires indépendants, comme le Haut Conseil des finances publiques, signalent que ces règles n'ont pas été respectées. De ce point de vue, l'élargissement des compétences du Haut Conseil est, à notre sens, utile et bienvenu. Mais les lois de programmation et les règles budgétaires seront toujours relativement faciles à contourner et leur non-respect sera difficile à sanctionner efficacement : nous pourrons toujours souverainement décider de ne pas appliquer ce que nous avons précédemment voté. Bref, comme le disait souvent Philippe Séguin lorsqu'il présidait la Cour des comptes, la volonté politique est bien plus importante que les règles budgétaires. Elle devra être très forte pour assainir nos comptes publics et réduire durablement les dépenses publiques.

profonde, allant au-delà des contingences de la période. Je m'en expliquerai en axant mon propos plus spécialement sur les collectivités territoriales, ainsi que l'a indiqué Christine Lavarde.

l'introduction de nouveaux objectifs pluriannuels dans la loi de programmation, ainsi que son extension à cinq ans et la fusion des débats d'orientation des finances publiques et sur le programme de stabilité, obéit à une logique attendue. Les corrections sémantiques et la clarification de certaines procédures ou présentations sont les bienvenues, qu'il s'agisse des affectations de taxes et de fonds de concours, de la mise en oeuvre d'un compteur des écarts constatés ou encore de la faculté de réviser les trajectoires. territoriales », je suis nécessairement sensible au nouveau traitement des prélèvements sur recettes et au recentrage sur leurs effets en termes de péréquation. De même, je salue le nouveau rapport annexé au projet de loi de finances, qui pourra constituer le support d'un débat sur l'ensemble des finances locales.

locales (CFL) seront très loin de jouer ce rôle. Certes, nous ne sommes pas un État fédéral ; mais pourra-t-on encore longtemps différer la réflexion qu'appellent la substitution des impôts nationaux à des impôts territorialisés et le besoin d'une péréquation verticale, autre que celle qui est appliquée au sein de l'enveloppe normée ?

relèverait de cette exigence, alors que nous poursuivons ce déphasage entre deux écosystèmes qui coexistent, sans dialogue réel, dans une impasse institutionnelle et démocratique entre le national et le local.

appliquer pendant cinq ans, en tenant compte de la conjoncture économique, des besoins différenciés, des nécessités sectorielles, du contexte international, des opérations militaires, et j'en passe. Or, depuis 2008 et la loi de programmation des finances publiques pour

n'a formalisé la doctrine des principes budgétaires. En effet, ils n'avaient pas comme principal souci la notion d'équilibre. Sous prétexte de résorber la dette publique, érigée en problème économique fondamental, ce texte crée une

commission ? M. Savoldelli vient de le dire, il demande ni plus ni moins que la suppression de l'article 1. Or cela aurait pour effet de maintenir en l'état le droit existant, ce qui n'est pas non plus

à la programmation et à la gouvernance des finances publiques procèdent, comme vous le savez, d'obligations européennes résultant du

Vous le savez, à droit constitutionnel constant, le Gouvernement ne peut pas être contraint juridiquement de proposer la révision d'une loi de programmation des finances publiques, alors même-

deux catégories de lois de programmation des finances publiques : les lois de programmation initiales et les lois de programmation rectificatives. rectificatives. Si les lois de programmation initiales doivent prévoir l'ensemble des éléments que les dispositions organiques regardent comme relevant du domaine obligatoire, les lois de programmation rectificatives pourront se limiter, elles,

que le solde public ne peut constituer, en soi, une boussole pour les choix budgétaires que nous voudrions opérer. M. Franck Waserman, professeur de droit public, explique d'ailleurs très bien le caractère tout à fait illusoire de la notion d'équilibre : « L'équilibre L'équilibre apparaît davantage comme un paramètre économique, voire pour certains, un objectif, que comme un principe structurant qui puisse se couler dans les formes du droit. C'est sans doute une des raisons pour lesquelles l'équilibre n'a jamais été formalisé comme un principe juridique des finances publiques, et qu'il n'a probablement pas vocation à l'être un jour. donc oublier l'idée selon laquelle les finances publiques doivent être nécessairement équilibrées et considérer les enjeux et les urgences- climatiques, sociales et environnementales supprimer les références aux traités européens et à leurs indicateurs, tels que « l'effort structurel »- défini à l'article 1 comme « l'incidence des mesures nouvelles sur les recettes et la contribution des dépenses à l'évolution du solde structurel les mécanismes de correction et autres contraintes européennes pesant sur les grandes orientations de la politique économique et budgétaire de la France. La logique qui les sous-tend est tout à fait symptomatique de la suprématie de la sphère européenne et de ses dogmes sur les intérêts nationaux. Ces multiples références et le fait de calquer nos finances publiques

soulignait ainsi que la trajectoire de solde structurel de la loi de programmation 2018-2022 s'écartait des engagements européens de la France, en retenant une réduction du déficit structurel « inférieure au minimum requis par les règles européennes Nous proposons donc au contraire que les lois de programmation déterminent une planification traduisant les besoins de la Nation, et concourent à l'application des principes sociaux, économiques et environnementaux définis dans la Constitution, le préambule de la Constitution de 1946 et la Charte de l'environnement

En conséquence, nous ne considérons pas comme souhaitable l'objectif d'évolution des recettes, car il constituerait une forme d'objectif concurrent, qui créerait de la confusion dans ce pilotage budgétaire. Nous proposons donc de revenir à la rédaction du texte adoptée

satisfait pas. Nous sommes sous la tutelle des institutions européennes, au premier rang desquelles la Commission ! Le traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire, signé en 2012, impose bien à vingt-deux États, dont le nôtre,

puis en 2011 -que la règle d'équilibre structurel et le mécanisme de correction « prennent effet dans le droit national des parties contractantes au moyen de dispositions contraignantes et permanentes, de préférence constitutionnelles, ou dont le plein respect et la stricte observance tout au long des processus budgétaires nationaux sont garantis de quelque autre façon.

reprise économique durable. Ce verrou doit sauter. En attendant ce changement, un élargissement des objectifs de la programmation des finances publiques s'avère nécessaire et potentiellement fructueux. l'objectif de l'équilibre budgétaire repose sur l'unique indicateur du PIB. Or ce dernier est non seulement décorrélé du bien-être de la population, mais il est lié également à l'augmentation de la pollution. Nous proposons donc qu'il soit compensé par un autre indicateur. Cet amendement vise ainsi à introduire un critère qualitatif

Même avis. À nos yeux, l'article 34 de la Constitution limite les considérations de la loi de programmation des finances publiques à des trajectoires budgétaires et à des indices économiques. Pour cette raison, le Gouvernement

M. Didier Rambaud. Cet amendement vise à revenir à la rédaction de l'Assemblée nationale concernant l'objectif d'évolution de la dépense des administrations publiques, en supprimant la référence aux « dépenses d'avenir L'objectif d'évolution des dépenses des administrations publiques introduit par ce texte est un outil comptable de suivi et de pilotage des finances publiques. Il n'a donc, par nature, pas vocation à distinguer les dépenses d'avenir et les dépenses de fonctionnement, à présenter une vision consolidée de l'évolution des dépenses par rapport à la programmation. Comme je l'ai souligné lors de la discussion générale, nous avons la possibilité de doter la LOLF de nouveaux outils performants. J'ose espérer qu'il puisse être question d'outils neutres et transpartisans.

C'est un indicateur, non normatif, qui exprime politiquement l'intention du législateur en matière d'évolution des dépenses. La notion de « dépenses d'avenir » est, comme vous le dites, difficile à cerner de manière précise. Nous avons eu, vous le savez, ce débat en commission. C'est la raison pour laquelle la commission des finances propose que ces dépenses et les choix méthodologiques du Gouvernement soient explicités dans le rapport annexé à la loi de programmation

dans cet hémicycle. L'Observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion sociale a produit en 2015 une étude visant à déterminer quels étaient les besoins minimaux des personnes pour participer effectivement à la vie sociale. Alors que chaque poste de dépense a été passé au crible, il est apparu que, selon une multiplicité de variables, notamment le lieu et le type d'habitation, ainsi que le nombre de personnes composant le ménage, les besoins minimaux oscillaient entre 1 424 euros et 3 284 euros. Si vous tenez absolument à plafonner les dépenses, pourquoi ne pas déterminer leur niveau minimal ? Ce serait tout à fait conforme aux objectifs de la programmation pluriannuelle des finances publiques, qui vise à prévoir à long terme les besoins essentiels de la Nation.

Doit-il être fort ou faible ? Mais où est la force et où est la faiblesse dans les circonstances actuelles ? La crise que nous vivons est une crise de la société dans l'État, la crise d'une société façonnée par l'État et délaissée par l'État sous la V République. Elle nous apprend qu'il y a deux choses que l'on ne saurait abolir : d'un côté, les besoins élémentaires de chacun et chacune des membres de la société ; de l'autre, les besoins de l'État requis pour les satisfaire. C'est dans cette double impossibilité ou dans cette double résilience qu'il faut, nous semble-t-il, essayer de réfléchir à nouveau à l'État,

Dans la mesure où ces dispositions sont purement programmatiques, la présentation proposée renforce l'information du Parlement sur les intentions du Gouvernement, ce qui est bienvenu.

Toutefois, sa déclinaison par sous-objectifs sur cinq ans, comme vous le proposez, nous apparaît plus complexe compte tenu des caractéristiques propres de chaque sous-objectif, notamment des déterminants de leur évolution.

M. Éric Bocquet. Nous voulons borner la durée d'une loi de programmation des finances publiques à celle du mandat des députés à l'Assemblée nationale. C'est une question de cohérence. La rédaction actuelle précise seulement une condition minimale de durée de programmation de trois ans, ce qui nous paraît insuffisant. il apparaît qu'une telle rédaction pourrait avoir pour conséquence un artifice à nos yeux inutile, car le prochain gouvernement pourrait déposer un projet de loi de programmation des finances publiques en 2025 ou, pis encore, en 2026. La programmation ainsi soumise à examen se révélerait être un simple artifice de communication. Il est assez évident que la programmation serait remise en cause par l'avènement d'une nouvelle majorité, car c'est le jeu démocratique. Même dans la perspective d'une révision à la suite d'une crise, par exemple sanitaire, ayant rendu caduque la précédente programmation, il paraît inopérant d'engager le mandat suivant. Même dans l'hypothèse d'une majorité reconduite d'un mandat législatif à l'autre, un projet de loi de programmation pourrait tout à fait être débattu et permettrait, de la sorte, d'affiner les principaux indicateurs constituant le socle des prévisions adossé à la programmation. nous considérons que les lois de programmation pourraient, conformément à l'article L.O. 121 du code électoral, ne pas perdurer au-delà du troisième mardi de juin de la cinquième année qui suit l'élection de l'Assemblée nationale.

? L'article 5 de la loi organique du 17 décembre 2012 relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques prévoit effectivement qu'un rapport est annexé à la loi de programmation et qu'il fait l'objet d'une approbation.

dans la mesure où le législateur organique n'est pas habilité par la Constitution à prévoir les modalités de vote des dispositions des lois de programmation, contrairement à la situation qui prévaut s'agissant des lois de finances et du financement de la sécurité sociale. La commission demande donc le retrait de cet amendement.

Mme Isabelle Briquet. Par le biais de la création d'un article 1 E de la LOLF, le présent article introduit une annexe visant à éclairer le Parlement sur la situation macroéconomique et financière du pays. du pays. Notre amendement a pour objet d'insérer dans ce rapport une présentation des fourchettes haute, moyenne et basse des évolutions attendues des taux d'intérêt et de leur impact sur les finances publiques. il s'agit d'un élément important pour jauger de la crédibilité de la trajectoire budgétaire pluriannuelle retenue par le Gouvernement. Et nous n'en disposons pas actuellement. Ces fourchettes auraient incontestablement une utilité pour évaluer la stratégie budgétaire du Gouvernement et pour préciser les prévisions budgétaires sur lesquelles sont fondés les projets de loi de finances et de finances rectificative.

Cet amendement vise à renforcer la clarté du débat parlementaire et la lisibilité de la loi de programmation des finances publiques.

en matière d'évolution du solde, des dépenses, des recettes et de l'endettement, et, d'autre part, les dispositions normatives afférentes à la gestion des finances publiques et à l'information du Parlement. On améliorera ainsi la présentation de la loi de programmation.

l'évaluation à moyen terme des ressources de l'État, ainsi que de ses charges ventilées par grandes fonctions, et, d'autre part, la liste des missions, des programmes et des indicateurs de performances associés à chacun de ces programmes, envisagés pour le projet de loi de finances de l'année suivante.

Ces délais marquent le joug des institutions européennes sur notre calendrier budgétaire ; ils attestent du peu de considération pour le temps dont le Parlement bénéficie pour examiner ce document structurant de la politique nationale. Au demeurant, aucune remarque formulée pendant les débats ne pourrait être transcrite dans le document transmis à la Commission européenne.

la Constitution, avait fait devant le Sénat une déclaration portant sur le projet de programme de stabilité 2014-2017. C'est une pratique tout à fait indispensable, qui permet d'échanger des visions politiques et de marquer, ne serait-ce que symboliquement, des différences de vision sur la politique nationale et sur la conception à long terme des finances publiques. l'avis de la commission ? Cet amendement a pour objet que le débat organisé sur le programme de stabilité et le rapport d'orientation des finances publiques soit suivi d'un vote.

européenne, le projet de programme de stabilité. Le Parlement débat de ce projet et se prononce par un vote. » L'article 48 de la LOLF, qui vise l'actuel rapport d'orientation des finances publiques, ne prévoit pas

En pratique, cet amendement n'aurait pas les effets recherchés par ses auteurs. Toutefois, il me paraît utile de demander au Gouvernement s'il souhaite, à l'avenir, que le débat sur le programme de stabilité et sur le rapport d'orientation des finances publiques soit suivi d'un vote. l'avis du Gouvernement

Le scrutin est ouvert.

d'euros. La moitié des emplois de cette ressource en 2020 aurait donc toujours échappé à la connaissance des parlementaires. En outre, cette information est laconique, comme pour les décrets d'avance. de ces raisons, nous demandons la suppression de l'article 4 A et, plus généralement, l'abolition de cette pratique qui crée plus de nuisances pour notre démocratie budgétaire qu'elle n'est utile à la société. D'autres solutions existent pour satisfaire les besoins de crédit dans l'urgence. Quel

L'Assemblée nationale souffre énormément du raccourcissement des délais. Le Gouvernement ne peut se prévaloir de l'article 47 de la Constitution pour justifier de tels resserrements du calendrier. L'année précédente fut marquée par un regrettable record : les

soit, nous comprenons tous que ce ne sont pas là des délais convenables pour préparer le travail en commission. De façon à éviter des dysfonctionnements préjudiciables à la démocratie et à la qualité des débats budgétaires, nous proposons d'inscrire dans la loi un délai incompressible de dix jours entre le dépôt du PLF et son examen en commission.

Ce que nous voulons, c'est aussi inverser les saisons ; moins d'automne de l'autorisation, plus de printemps de l'évaluation. Nous voulons éviter d'alourdir encore le dispositif d'autorisation parlementaire qui a lieu à l'automne, ce qui risque de produire des commissions élargies ou un vote pour chaque programme budgétaire ; nous préférons renforcer l'évaluation du printemps ».

nous pensons qu'il faut au contraire renforcer l'autorisation parlementaire, même dans des circonstances exceptionnelles. Nous demandons de pouvoir voter sur les programmes, afin d'adopter des positions plus fines, plus précises, pour ne pas avoir à rejeter en bloc des crédits auxquels nous pourrions souscrire. Lors de la dernière loi de finances, il nous était seulement possible de voter pour ou contre le plan de relance ou de nous abstenir ; trois choix pour prendre position sur 36,2 milliards d'euros d'autorisations d'engagement sur une année

Notre amendement a été déclaré irrecevable au titre de l'article 40, que nous essayons d'infléchir en modifiant sa transcription dans la LOLF. Tout cela est logique. D'ailleurs, on dit souvent que les lois de la logique ne peuvent être violées que par ceux qui les possèdent ... Nous essayons donc de nous en vue de nous opposer à l'article 40 de la Constitution, bien que les deux auteurs de cette proposition ne soient pas d'accord au sujet de cet amendement. Laurent Saint-Martin a renvoyé à un autre texte le soin de débattre de cette question.

Elle est disponible au format électronique en données ouvertes. À partir de ce document, il n'est pas très difficile de déduire le montant des crédits non consommés. Je le précise, un amendement de la commission prévoit de renforcer l'obligation de publier ces données

au budget de l'État, ainsi qu'à l'ensemble des collectivités locales, n'est pas tout à fait adaptée à la situation que nous vivons aujourd'hui.

il se trouve que la définition de ces dépenses, notamment d'investissement, qu'il s'agisse d'immobilisations corporelles ou incorporelles, ne paraît pas pertinente dans la mesure où elle n'inclut que des dépenses visant à accroître l'actif de l'État, alors que certaines dépenses de fonctionnement visent à à accroître l'actif de la société d'une manière plus générale. En effet, face aux enjeux que je viens d'évoquer, la puissance publique doit aujourd'hui à la fois investir dans le capital humain et assumer des dépenses, lesquelles, dans la nomenclature comptable actuelle, sont considérées comme des dépenses de fonctionnement, alors qu'elles sont nécessaires pour oeuvrer à la transition écologique. L'urgence climatique oblige les gouvernements à agir très rapidement au regard des enjeux et de l'accélération brutale

relayée par les acteurs privés, pourrait entraîner à échéance rapide, soit en 2030, une perte de PIB de l'ordre de 10 %, ce qui aurait bien évidemment des conséquences sur les équilibres budgétaires à venir. est donc urgent de revoir cette nomenclature comptable, pour prendre en compte la solvabilité à venir de l'État au regard des enjeux climatiques qui sont devant nous.

retirer votre amendement.

du Gouvernement ? Le Gouvernement considère que cet amendement va un peu plus loin qu'une clarification rédactionnelle, puisqu'il tend à alléger l'encadrement des prélèvements sur recettes, les PSR, en supprimant les conditions de définition et d'évaluation de leur destination

le ministre délégué. J'ai indiqué dans la discussion générale que j'aurai l'occasion de présenter un amendement visant à restreindre quelque peu le champ du rapport sur les finances locales. cet amendement, il s'agit de ne pas faire figurer dans le rapport l'examen de l'évolution des charges résultant des transferts de compétences entre l'État et les collectivités. En effet, dès lors que la collectivité se voit transférer la responsabilité d'une compétence, elle est aussi responsable des moyens qu'elle y consacre, après avoir perçu les allocations de compensation telles que calculées logiquement. L'évolution des charges transférées ne dépend plus que des décisions prises par la collectivité et des modalités de gestion qu'elle a choisies. C'est la raison pour laquelle nous proposons de supprimer l'alinéa qui définit le contenu du rapport sur les finances locales.

dans le cadre du sondage d'Odoxa-Backbone Consulting pour France Info et Le Figaro de mai 2019, six Français sur dix plébiscitent un maintien ou une hausse du nombre d'agents, contrairement à la promesse de campagne d'Emmanuel Macron de réduire de 120 000 le nombre de postes de fonctionnaires sur le quinquennat.

d'une disposition avant tout technique, puisque la notion d'autorisation d'engagement est pertinente pour les dépenses portant sur des projets spécifiques ayant une durée supérieure à une année. Telles sont les raisons pour lesquelles j'émets un avis défavorable

nous pensons que les reports de crédits constituent le meilleur outil de gestion, seul à même de garantir une véritable pluriannualité des dépenses publiques. Si nous pouvons discuter des pourcentages, nous proposons que soit ramené à 5 % le montant des autorisations d'engagement pouvant être reportées par programme, alors qu'il n'existe aujourd'hui aucune limite, et à 1 % pour le montant des crédits de paiement. Les majorations pourraient être autorisées dans le cadre d'une loi de finances rectificative, tous titres confondus indistinctement, selon que ce sont des dépenses de personnels ou des dépenses sur d'autres titres, dans la limite actuelle de 3 %. Aujourd'hui, l'outil nécessaire que constituent les reports de crédits a été dévoyé au profit d'effets d'annonce, rendant insincères les lois de finances que nous votons. L'épisode de l'année dernière, même en période de crise, est extrêmement préoccupant de ce point de vue. Ainsi, des crédits de 31,6 milliards d'euros, soit 8,3 % des dépenses nettes du budget général,

La sous-consommation des crédits en fin d'année reflète, au-delà des incertitudes liées à la crise sanitaire, un manque de réalisme des prévisions budgétaires.

sous le contrôle efficace des deux rapporteurs. Nous avons précisé que les budgets annexes peuvent retracer les dépenses associées à celles qui étaient déjà retracées dans la LOLF. C'est un élargissement qui nous permet de nous rapprocher de la pratique.

Il existe donc un besoin manifeste de disposer d'informations plus précises et exhaustives pour évaluer la performance de l'action de l'État actionnaire dans la gestion de ses intérêts patrimoniaux. Quel est l'avis de la commission

du compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État », d'établir à l'aune de quelle distinction un tel partage en sections serait réalisé. En l'occurrence, les différentes dépenses réalisées par l'APE sur le programme 731, qu'il s'agisse d'augmentations de capital, de l'octroi de prêts d'actionnaires, d'investissements financiers de nature patrimoniale, ne sauraient être individuellement attachées par nature à certains types de recettes versées sur le CAS, notamment les produits de cessions, les récupérations de dotations en capital, les dotations du budget général ou encore les remboursements de créances. Instaurer une telle séparation d'affichage entre les deux sections du CAS n'est donc pas compatible avec les conditions réelles d'exécution du compte. Je ne doute pas que nous puissions améliorer,

Cet amendement vise à renforcer l'information du Parlement en cas de mobilisation de crédits exceptionnels au titre des participations financières de l'État

Le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État » fait toutefois exception à ce principe. Si la pratique a prouvé l'utilité de cette dérogation, elle a également souligné la nécessité de l'assortir d'un pouvoir d'information du Parlement. C'est la raison pour laquelle nous proposons que, en cas de versement du budget général excédant le plafond de 10 % des crédits initiaux du compte d'affectation spéciale «

avec une information aussi fidèle qu'exhaustive du Parlement. L'information préalable proposée par MM. les rapporteurs n'apporterait pas véritablement de valeur ajoutée.

que soit averti également le président ou la présidente de la commission des affaires économiques, car il s'agit de mettre de l'argent public dans des entreprises qui relèvent,

Par exemple, donc, la quatrième loi de finances rectificative pour 2020 a instauré des avances remboursables destinées à soutenir les autorités organisatrices de la mobilité (AOM) pour faire face aux conséquences de l'épidémie de covid-19. Le remboursement de ces avances

considérant que le Parlement devait donner son avis sur le montant des sommes demandées aux étudiants, avait voté contre cet article 48. À l'Assemblée nationale, plusieurs députés avaient dénoncé « un empiétement de l'exécutif sur le législatif

Le Conseil constitutionnel, en 2019, a considéré, sur le fondement du treizième alinéa du préambule de la Constitution de 1946, que l'exigence constitutionnelle de gratuité de l'enseignement s'appliquait aussi à l'enseignement supérieur public.

de la loi budgétaire, la possibilité de débattre aussi de ces droits d'inscription dont la nature s'apparente à celle de la CVEC. Bravo ! Quel est Monsieur le sénateur Ouzoulias, par votre démonstration, vous venez de rappeler que, aujourd'hui, les droits d'inscription à l'université sont fixés par arrêté. Votre proposition pose des problèmes de principe : problème de séparation entre la loi et le règlement,

alors que leur nature exacte, redevance pour service rendu ou taxe affectée aux universités, vous l'avez dit, continue de faire l'objet d'un débat juridique. En tout état de cause, une ressource de l'État ne fait pas partie du domaine obligatoire des lois de finances

l'avis du Gouvernement ? Même avis. Monsieur Ouzoulias, J'ai compris que vous n'étiez pas insensible à mon argument : il faudra que nous nous posions la question de savoir pourquoi ce que je considère comme une taxe fait l'objet d'un autre traitement, dans le cadre de la loi budgétaire, que la CVEC, qui est également une taxe affectée

Mme Raymonde Poncet Monge. Les indicateurs de performance constituent l'outil central de l'évaluation de la dépense publique. Pourtant, cet outil néglige les conséquences environnementales de la dépense publique. Comme l'illustre la décision du 1 juillet 2021 du Conseil d'État, les efforts de la France sont largement insuffisants pour atteindre l'objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre fixé pour 2030. Les modalités d'élaboration et d'évaluation du budget de l'État ont leur part de responsabilité dans cette situation.

En effet, la conception même du budget vert conduit à une impasse : toute dépense permettant une amélioration par rapport à l'existant est considérée comme favorable à l'environnement, même si cette amélioration est minime et insuffisante pour atteindre les engagements internationaux de la France. En outre, et à l'inverse, les dépenses pour lesquelles les informations nécessaires à la détermination de leur impact environnemental ne sont pas disponibles sont arbitrairement jugées neutres. Face aux biais inhérents au budget vert, il est nécessaire de mobiliser les indicateurs de performance en faveur de la protection de l'environnement. Les cinq indicateurs choisis- économie circulaire et déchets, gestion de la ressource en eau, lutte contre le réchauffement climatique, lutte contre les pollutions, biodiversité et protection des espaces naturels

tout à fait louable, de permettre à une loi de finances de comporter des dispositions autorisant le transfert de données fiscales lorsque celui-ci a pour effet de limiter les charges ou d'accroître les ressources de l'État.

visait à ajouter l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) aux organismes qui peuvent obtenir, « sur demande ou d'office, tout élément recueilli au cours d'une instance civile ou d'une information criminelle ou correctionnelle, y compris lorsque celle-ci s'est terminée par un non-lieu, de nature à faire suspecter le caractère frauduleux d'une demande d'asile. » L'objectif était simple et posé par l'auteur de l'amendement dont était issue cette disposition, M. Laurent Saint-Martin : interrompre, le cas échéant, le versement de l'allocation pour demandeur d'asile en cas de fraude à la demande d'asile. Même Mme Schiappa avait considéré cette disposition comme « juridiquement discutable, voire contestable, dans la mesure où elle donne la possibilité à l'OFII d'accéder à des données extérieures aux champs légaux de ses missions. Nous nous étions opposés avec force à cette disposition, mais ce n'était qu'un article noyé parmi d'autres, sans étude d'impact, introduit par amendement ; les conditions de travail, complexes, n'avaient pas permis de se mobiliser contre un dispositif aussi contestable, soulevant d'ailleurs plus de questions qu'il ne résout de problèmes, donnant lieu à des risques sociaux majeurs pour les demandeurs d'asile, dont chaque passage au tribunal, même s'ils en sortent innocentés, pourrait engendrer des conséquences néfastes.

À ce stade, il me paraît utile que le Gouvernement nous indique quelle serait l'importance, notamment sur le plan budgétaire, des transferts de données qu'il pourrait être amené à demander. Quel est l'avis du Gouvernement

L'application de l'alinéa 24 de l'article 5 permettrait d'inclure dans une loi de finances ce type de dispositions destinées à des administrations de l'État gérant des dispositifs d'aide ou de subvention subordonnés à des conditions de ressources. Grâce à une telle communication, ces administrations de refuser une aide avant son octroi ou de retirer une aide indûment accordée pour sauvegarder les ressources de l'État. La DGFiP a développé des échanges informatisés qui permettent de réduire les coûts de gestion. Notre objectif n'est pas